Concrètement, cette absence de compensation entraînerait de lourdes difficultés financières pour ces structures et une diminution de leurs actions de prévention, d’accueil, d’écoute et d’accompagnement juridique des femmes victimes de violences, avec à la clé des fermetures et des licenciements. Le présent amendement vise à remédier à cette situation, qui serait particulièrement regrettable pour la prise en charge des femmes victimes de violences sur tout le territoire, en renforçant les crédits du programme 137, « Égalité entre les femmes et les hommes », à hauteur de 7 millions d’euros. La parole

assise financière suffisante pour l’absorber. Outre un moindre accompagnement des femmes victimes de violences, nous craignons la fermeture de certains lieux d’accueil et le licenciement de leurs salariés. Le présent amendement, que nous sommes nombreux à défendre, vise donc à transférer 7 millions d’euros du programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », au programme 137, « Égalité entre les femmes et les hommes ». Nous demandons bien sûr au Gouvernement de lever le gage sur

d’accompagnement des victimes de violences. Comme cela a déjà été dit, cette absence de compensation financière risque de mettre ces associations dans une situation économique particulièrement critique. Elles devraient faire face à des difficultés majeures, qui pourraient compromettre les missions essentielles que sont la prévention, l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des femmes victimes de violences, ainsi que le soutien juridique.

Il est indispensable de garantir la pérennité et la viabilité de ces associations, afin qu’elles puissent continuer à accompagner efficacement ces femmes partout en France. Le Gouvernement a déjà fait des pas importants pour aider les femmes dans la détresse, mais cette lutte sera vaine si nous affaiblissons les associations qui leur apportent une aide cruciale et parfois même vitale. Pourtant, en l’absence de compensation financière pour le versement de la prime Ségur, qui est obligatoire depuis le 6 août dernier, ces associations doivent déjà réduire leurs services, geler leurs recrutements, voire recourir à des licenciements économiques.

Les centres d’information sur les droits des femmes et des familles exercent la mission d’intérêt général qui leur est confiée par l’État, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale,

l’État a répondu favorablement à une demande, formulée de longue date par le secteur associatif et médico social, de revalorisation des salaires. Cette mesure était nécessaire dans un secteur où les salariés, en très grande majorité des femmes, exercent des métiers difficiles et mal rémunérés. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une participation de l’État au financement de la prime Ségur versée par les centres de protection maternelle

aux salariés du secteur sanitaire, social et médico social privé ne peut se faire sans compensation financière de la part de l’État, et souligner la non prise en compte de ce problème dans le projet de loi de finances pour 2025. Aussi, le transfert symbolique d’un million d’euros que nous proposons vise non pas à amoindrir l’enveloppe prévue pour financer la prime Ségur dans les centres de protection maternelle et infantile, mais à interpeller le Gouvernement sur le besoin d’une prise en charge financière pour la mise en œuvre de cette mesure dans les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes de violences. Il y va de l’avenir de ces associations, qui jouent un rôle essentiel et indispensable en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. C’est le cas des CIDFF, qui nous ont fait part de leurs grandes difficultés financières pour l’année à venir. Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la Lolf, il est proposé de compenser cette dépense par le transfert de 1 million d’euros depuis l’action n° 17, « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables », du programme 304,

Le 5 août 2024, le Gouvernement a acté l’extension de cette prime aux salariés du secteur sanitaire, social et médico social privé relevant de la convention

l’apparition de véritables zones blanches dans l’accès aux droits, ce qui sera particulièrement préjudiciable pour les femmes et les publics les plus vulnérables. Concrètement, certaines associations seront contraintes de licencier, voire de cesser leur activité faute de fonds propres suffisants pour mettre

Corinne Féret. Cet amendement vise à favoriser le développement territorial des solutions temporaires de répit partagé, destinées à accompagner les aidants et leurs proches en situation de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge. Ces résidences de répit, qui sont cofinancées par les départements et l’État, nécessitent un engagement fort et ciblé de la part de l’État, notamment les crédits de cette mission budgétaire. Je rappelle que nos résidences de répit partagé proposent l’accueil temporaire à vocation médico sociale de la personne aidée, en présence d’un ou plusieurs aidants familiaux, qui bénéficient conjointement d’une offre de tourisme et de vacances adaptées à leurs attentes et à leurs besoins réciproques. C’est vraiment tout à fait spécifique.

Toutefois, je me souviens que l’an dernier, la ministre au banc avait assuré à nos collègues qu’au moins cinq plateformes de répit partagé seraient ouvertes d’ici à 2027, dont une dans les Landes. Peut être peut elle nous préciser où en est la mise en œuvre de cet engagement

Mme Raymonde Poncet Monge. La nette sous insertion professionnelle des personnes malvoyantes est due à de nombreux facteurs, inhérents aux discriminations validistes encore omniprésentes sur le marché du travail et dans notre société,

Par cet amendement, nous appelons à développer l’accès aux aides et aux services à destination des personnes malvoyantes en luttant contre le non recours aux aides et en augmentant les moyens alloués aux prestations d’appui spécifiques (PAS).

Les épiceries sociales et solidaires doivent faire face à de nombreux défis. L’inflation sur les produits alimentaires a atteint 20 % en deux ans. De nombreuses épiceries sociales et solidaires ont dû refuser d’accueillir de nouvelles personnes.

de la subvention a beaucoup diminué du fait de l’inflation. L’an dernier, le Sénat avait déjà soutenu ces demandes. Il nous paraît nécessaire de tenir compte de l’évolution du nombre de structures et de bénéficiaires, mais aussi de

Mme Raymonde Poncet Monge. L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales est déployée sur tout le territoire depuis le 1 décembre 2023. Cependant, à ce jour,

des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, vise à créer un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de cette aide universelle d’urgence dans la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », dont elle dépend. En effet, la communication de cet indicateur devrait être régulière, afin d’alimenter le débat public, ainsi que le travail parlementaire lors de la préparation de chaque budget. Il s’agit de mesurer l’impact de ce dispositif.

dans les crédits que vous venez de voter pour accompagner les communes dans leurs nouvelles compétences liées au déploiement du service public de la petite enfance. Cet amendement vise à donner une base légale à l’État pour la bonne délégation de ces crédits,

celle là même qui bénéficie aux communes les plus petites. Notre pays compte 25 000 communes de moins de 1 000 habitants, qui ont besoin d’être bien plus accompagnés qu’elles ne le sont aujourd’hui pour traiter la question du zéro artificialisation nette (ZAN) ou celle de la transition énergétique.

vise à accompagner certains territoires dans leur stratégie de sobriété foncière au regard des enjeux liés à l’artificialisation des sols et à l’étalement urbain. Elle aide des collectivités territoriales dans la définition de leur stratégie urbaine, pour réinventer un modèle de densification ou de dédensification, en s’appuyant sur la qualité de vie qu’offre une ville à taille humaine. Ce programme a connu de vrais succès et permis à de nombreux territoires de régénérer

Nombre d’élus se sont engagés dans cette démarche, mais ils ont besoin d’un accompagnement. Or aucune réponse concrète n’est aujourd’hui apportée par le Gouvernement pour aider les communes à réussir cette mise en œuvre. La reconquête du bâti des centres bourgs et des centres de villages est un enjeu majeur.

d’expérimenter une aide aux maires ruraux pour des opérations dédiées à la réhabilitation, à la rénovation ou à l’adaptation de l’habitat, ainsi qu’aux opérations de reconversion du bâti en logements destinés à la location à prix maîtrisé ou à l’accession sociale à la propriété des habitants de ces mêmes territoires.

pour les agents de la fonction publique exerçant dans certaines communes de l’Ain et de la Haute Savoie, donc à proximité de la frontière suisse. Cette prime de résidence, égale à 3 % de leur traitement indiciaire, a vocation à permettre aux agents concernés de faire face aux tensions très fortes sur le marché immobilier local en raison de la proximité de l’agglomération de Genève. Le nord lorrain, en proie, lui aussi, à des tensions importantes sur le marché de l’immobilier local, en raison de sa proximité géographique avec le Luxembourg, ne fait pas l’objet de mesures d’accompagnement de ses agents. Dans un souci d’équité, cet amendement vise au versement d’une prime identique pour les agents des communes frontalières du Nord lorrain.

Poursuivre cette politique publique de soutien, avec des montants raisonnables au regard de la valeur sociétale apportée sur les territoires, répond à un objectif d’efficacité de la dépense publique et de cohérence de l’action menée.

Nous pensons qu’il faut réabonder ces crédits à hauteur de 10,5 millions d’euros. Afin de ne pas faire

pour la période 2021 2027. Cette mesure répond à une nécessité impérieuse de santé publique et de justice environnementale aux Antilles. En effet, le chlordécone a entraîné une contamination durable des sols et des eaux, affectant gravement la santé de nos populations locales. Une étude de Santé publique France de 2018 révèle que plus de 90 % des adultes en Guadeloupe et en Martinique présentent des traces de chlordécone dans leur organisme. Les conséquences sanitaires sont alarmantes, avec une incidence élevée de cancer de la prostate, reconnu comme maladie professionnelle liée à l’exposition au chlordécone. La persistance de ce polluant dans l’environnement, estimée à plusieurs siècles, nécessite des actions soutenues et financées de manière adéquate pour atténuer ces effets. Il est vrai que, en 2019, le gouvernement de l’époque avait débloqué une aide de 5,4 millions pour lutter contre cette pollution. Mais face à l’ampleur du problème, il est crucial de maintenir et de stabiliser ces financements à hauteur de 5 millions d’euros annuels pour les années à venir. Il nous faut renforcer les infrastructures de traitement de l’eau potable, soutenir les agriculteurs dans la transition des pratiques agricoles sûres et financer des programmes de dépistage et de prévention des maladies liées à l’exposition au chlordécone. Les deux amendements

à 1,5 milliard d’euros par an. La tarification incitative des déchets constitue un levier majeur d’amélioration, comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport du 27 septembre 2002. Or ce passage à la tarification incitative peut susciter des craintes parmi les ménages les plus modestes et les élus locaux, car il n’y a pas à ce jour de possibilité de définir une tarification sociale des déchets. Comme pour l’ensemble de la transition écologique, la fiscalité des déchets doit intégrer les principes de justice sociale pour être efficace. Les débats abondants en Dordogne, à la suite du passage du département en tarification incitative, montrent pourtant qu’une dimension sociale à la tarification des déchets est essentielle. En raison de l’opposition répétée ces dernières années de l’administration fiscale à la création d’une dimension sociale à cette tarification, le présent amendement vise à créer un un programme « Fonds de solidarité sociale, handicap et grand âge à la transition des territoires vers la tarification incitative des déchets », doté de 5 millions d’euros. En effet, le syndicat des déchets de la Dordogne indique que le besoin serait d’au moins 1 million d’euros.

cosignataire, vise à répondre au défi posé par la double insularité en Guadeloupe, en allouant 4 millions d’euros à la création d’un service public multimodal de transport maritime. La double insularité qui caractérise La Désirade, Marie Galante et Les Saintes aggrave les difficultés d’accès aux services publics, à l’emploi et à l’activité économique, tout en augmentant le coût de la vie pour les populations locales. Le financement proposé permettra de stabiliser juridiquement les obligations de service public dans les îles du Sud, assurant ainsi un transport régulier et accessible pour les passagers, les marchandises et les véhicules. En désenclavant ce territoire, il félicitera les échanges économiques, favorisera le développement du tourisme local et renforcera la cohésion sociale entre les différentes îles de l’archipel. Des initiatives similaires, en Corse ou dans d’autres territoires insulaires européens, ont montré l’efficacité de telles politiques pour réduire l’isolement géographique et stimuler l’économie locale. Voilà qui constitue un précédent solide pour soutenir une telle démarche en Guadeloupe. Quel est l’avis de

Loire, seulement 11 % de la masse d’eau est de bonne qualité. Cela justifie évidemment de reconduire les moyens budgétaires dédiés à la reconquête de la qualité de l’eau en Pays de la Loire, un programme spécifique

en Pays de la Loire

la contamination au plomb et au cadmium continue d’affecter la santé des familles riveraines du site et de polluer gravement les sols du territoire. Le 23 mai 2024, la cour d’appel de Douai a statué en faveur des cinquante et un requérants riverains de l’ancienne usine. Ces habitants subissent toujours les conséquences de cette contamination, même vingt ans après la fermeture. L’État, qui s’est pourvu en cassation, a toutefois laissé entendre, par le biais de la ministre Agnès Pannier Runacher, que les sommes correspondant à l’anonymisation des familles victimes leur seraient tout de même allouées. Cet amendement vise donc à verser la somme de 1,2 million d’euros, équivalente au montant total du préjudice reconnu pour les requérants.

équivalente des aides personnalisées au logement. Les forfaits de RLS, ainsi que les montants des ressources mensuelles maximales y ouvrant droit, sont revalorisés chaque année. Ces charges

1,1 milliard en 2025, afin de renforcer les fonds propres des bailleurs et de soutenir l’effort de construction et de rénovation. Aussi, cet amendement tend à modifier les règles d’indexation de certains paramètres de la RLS.

ou d’une délinquance locale, voire itinérante, qui cible les personnes vulnérables. Le préjudice pour les politiques publiques concernées est à la fois financier – les aides sont captées pour financer des travaux ou équipements mal réalisés ou défectueux – et réputationnel. Il conduit à la méfiance des ménages et nuit à l’image des entreprises du secteur, qui sont également victimes de la concurrence déloyale des écodélinquants. Dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, l’Ademe et l’Anah doivent avoir accès aux données des autres administrations. Les dispositions du présent amendement visent donc à lever les obstacles législatifs à la communication par les administrations à l’Ademe et à l’Anah d’éléments couverts par le secret professionnel

plus que les attaques cyber et la désinformation touchent l’ensemble du tissu économique et social, les institutions, les hôpitaux, les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les particuliers. La cyberguerre et les manipulations de l’information ont été largement documentées par la délégation parlementaire au renseignement que j’ai présidée jusqu’à récemment, ainsi que par la commission d’enquête sur les politiques publiques face aux opérations d’influences étrangères, présidée par mon collègue Dominique de Legge. La réduction des moyens du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) n’est donc pas cohérente. Pis,

L’IHEDN est aussi un centre de recherche de premier plan, qui alimente les débats publics et enrichit notre compréhension des enjeux contemporains de sécurité. En stabilisant son budget, nous lui permettons de maintenir ses missions à la hauteur des exigences. La parole est à M.

l’amendement n° II 1607. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », figurant à l’état B. Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

par avance, à sa future retraite d’ancien président de la République. Il deviendrait ainsi le premier président à renoncer au bénéfice de la loi du 3 avril 1955. En vertu de ce texte, qui est toujours en vigueur, les anciens chefs d’État se voient verser à vie, dès leur départ de l’Élysée, une pension équivalente au salaire d’un conseiller d’État, dont le montant n’est soumis à aucune condition d’âge, ni de durée de mandat, ni de revenus.

amendement vise à supprimer cette dotation, souvent assimilée à tort à une pension de retraite pour les présidents élus après le 1 avril 2022. Or les présidents de la République française ne bénéficient, pendant la période d’exercice de leur fonction, d’aucun

madame la ministre

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Son bon fonctionnement est indispensable à l’amélioration des connaissances et à l’émergence de solutions là où il s’agit de lutter contre les maladies animales ou de faire face à des impasses techniques résultant elles mêmes d’un déficit d’anticipation et d’orientation des priorités de recherche de la part des pouvoirs publics.

Mme la ministre.

le présent amendement vise à aller encore plus loin et à l’abaisser de 25 ETP supplémentaires pour le fixer à 325

l’entretien des 233 hippodromes français et l’organisation de 18 000 courses chaque année. Elle anime également 14 000 points de vente dans les territoires, où elle génère 29 000 emplois. L’autonomie de la filière hippique dépend à 93 % des revenus du pari hippique, lequel a aussi directement contribué aux recettes de l’État à hauteur de 825 millions d’euros. Or le nombre de parieurs a chuté de moitié au cours de la dernière décennie, passant de 7 millions

L’objectif d’éviter toute déstabilisation économique des filières en lien avec l’exploitation de jeux d’argent autorisés est inscrit dans la loi depuis 2010, à l’article L. 320 3 du code de la sécurité intérieure.

elle n’est plus à même de répondre aux nouveaux modes de consommation des joueurs, car ces modes ont évolué depuis 133 ans. Il faut conclure. D’ailleurs, dans son rapport de septembre 2023 dédié aux jeux d’argent, la Cour des comptes incite l’État à mettre en œuvre une vision d’avenir pour ce secteur

Pour rappel, ce dispositif finance des projets réalisés en France ou à l’étranger et considérés comme stratégiques pour l’économie française. Il peut s’agir, par exemple, de la construction et de l’exploitation d’usines de batteries de véhicules électriques, essentielles à la transition écologique. Nous proposons de sécuriser des projets industriels stratégiques sur le sol français en supprimant le critère d’exportation. En effet, depuis la mise en place du volet domestique de cette garantie en 2022, bien que tous les projets de réindustrialisation visent, à terme, des débouchés à l’international, la composante export peut intervenir à des stades différents du modèle d’affaires. Il apparaît donc nécessaire de ne pas conditionner l’octroi de la GPS à un critère d’export qui ne correspond pas systématiquement au niveau de maturité industrielle et commerciale des projets. Quel est l’avis de la commission ? Favorable.

au titre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles. Par ce mécanisme, il s’agit de soutenir les agriculteurs qui se trouvent dans une situation difficile du fait d’aléas climatiques, sanitaires

madame la présidente.

Compte tenu de la nécessité d’accélérer les actions en faveur de la transition écologique et énergétique comme de rendre compte aux citoyens de l’effort public déployé en la matière, il convient de franchir une nouvelle étape, en permettant aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants qui le souhaitent de mettre en place leur budget vert.

Son exposé des motifs se conclut explicitement sur l’enjeu financier qui préside à cette démarche gouvernementale. Les sommes en jeu pour l’État

amendement vise à modifier le régime de répartition de l’Ifer applicable en cas de renouvellement d’un parc éolien ou d’une installation photovoltaïque. Depuis la loi de finances pour 2019, les communes d’implantation d’un parc éolien

à la commune d’implantation une part minimale de 20 % de l’Ifer à l’occasion du renouvellement d’éoliennes installées avant le 1 janvier 2019 ou d’une installation photovoltaïque implantée avant le 1 janvier 2023 sur son territoire. Une telle mesure me paraît équitable et cohérente. Elle contribuera de plus à sécuriser les recettes locales, à renforcer l’acceptabilité des projets par

de créer une dérogation au secret professionnel au profit du Centre national de la musique (CNM). Cela permettra notamment de mieux contrôler les deux taxes qui financent l’activité de ce centre, la taxe dite et la taxe sur les spectacles vivants.

Dans le cadre du renforcement de notre aide publique au développement, nous devons veiller à ce que le cycle de reconstitution de cette association pour 2025 2028 bénéficie d’un fort soutien de la France.

pour les fonctionnaires qui sont en poste dans les outre mer. Nous souhaitons notamment offrir la possibilité aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires en activité à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, ainsi qu’à Wallis et Futuna,

été convoqué au sujet des retraites, je continue de dire qu’en la matière il faut garder les yeux ouverts : ce régime est un bon exemple d’une cotisation additionnelle obligatoire au bénéfice des fonctionnaires.

d’imposer une plus grande transparence des cabinets de conseil, conformément aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale. Si le Gouvernement a créé un jaune budgétaire dans le cadre du PLF pour 2023, ce document se révèle lacunaire et même décevant. En outre, les administrations persistent dans leur refus de publier les bons de commande et les livrables des consultants, malgré la jurisprudence de la

Madame Cukierman,

se livrent à une concurrence mondiale à l’aide de leurs outils d’influence, la création d’un tel document nous paraît essentielle aux fins d’analyser et d’améliorer nos politiques en la matière, d’autant que l’influence comme se caractérise comme couvrant un champ très large de politiques publiques relevant de ministères et d’opérateurs nombreux éducation, diplomatie, culture, attractivité commerciale, commerce extérieur, médias internationaux ou encore francophonie. Ce document permettra de rationaliser les données relatives à l’influence dans une source d’information unique, tout en présentant chaque année la stratégie mise en œuvre et les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. disposerons nous d’une meilleure visibilité sur l’effort financier consacré par l’État à cette politique, ainsi que sur les dispositifs mis en place pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente. Une analyse pourra être faite afin d’identifier les incohérences et d’éventuels doublons. L’élaboration de ce document par les administrations contribuera à améliorer l’information du Parlement sur la gestion des finances publiques et à conforter les démarches de pilotage et de décloisonnement largement engagées, garantes de l’efficacité de notre politique d’influence. Quel

visant à informer le Parlement sur l’impact des coupes budgétaires prises par décret en février 2024. Pour prendre un seul exemple, la mission « Aide publique au développement s’est vue délestée de plus de 700 millions d’euros ; il s’agit de la coupe budgétaire la plus importante réalisée lors de cette séquence de remise en cause de la loi de finances pour 2024.

au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les fonctionnaires d’État de La Réunion et de Mayotte. Je rappelle que, dans ces départements, la pauvreté touche plus particulièrement les personnes âgées et que ces populations perçoivent les pensions de retraite les plus faibles de nos régions et départements.

proximité de leur lieu de travail, notamment dans les zones frontalières. C’était il y a quelques jours, alors que nous examinions les crédits qui vont permettre la création d’une foncière de l’État : j’ai pris l’engagement que nous travaillions à créer des logements,

La séance est reprise. Nous allons procéder aux coordinations sur l’article liminaire et sur l’article d’équilibre. Je rappelle au Sénat que, aux termes de l’article 43, alinéa 3,